Monsieur le président,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

élu juge titulaire à la Cour de justice de la République le 21 octobre dernier, va être appelé à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l'article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.

Sans nier l'existence de deux sphères distinctes, nous ne pensons pas souhaitable de rigidifier les relations entre l'État et la sécurité sociale. Les assurés et les entreprises

grâce à un transfert très important de TVA. Près d'un quart du produit de la TVA est aujourd'hui affecté à la sécurité sociale, soit plus de 40 milliards d'euros. L'effort budgétaire qui est mobilisé à cet effet est d'une ampleur inédite. Alors que l'enveloppe prévue par la loi de finances rectificative du 30 juillet dernier s'élevait à 3,9 milliards d'euros, le coût du dispositif a été réévalué à un peu plus de 5 milliards d'euros. Compte tenu du coup projeté du second dispositif,

sociale (PLFSS) sur les exonérations de cotisations et leur compensation et, d'autre part, sur l'évolution ces dernières années des exonérations et exemptions de cotisations sociales. ont augmenté de 32,8 milliards d'euros entre 2013 et 2021, passant de 34 à 66 milliards d'euros, ce qui entraîne une disparition de cotisations sociales et une augmentation des compensations de l'État, et donc une fiscalisation de plus en plus forte de la sécurité sociale. En remettant en cause la loi Veil, c'est-à-dire en refusant de compenser intégralement les exonérations de cotisations sociales, l'État agit comme si la sécurité sociale était devenue son porte-monnaie, comme s'il pouvait agir comme bon lui semble. Non seulement les exonérations de cotisations sociales n'ont jamais démontré leur efficacité économique, mais leur compensation intégrale ou partielle par l'État fragilise notre modèle

nouvelle pression sur les hôpitaux. Ne pas compenser intégralement les exonérations, les exemptions et les allégements de cotisations revient à déstabiliser ce pilier qu'est la sécurité sociale. Je suis saisi

La contribution demandée aux organismes complémentaires d'assurance maladie s'applique sans différenciation aux mutuelles. Or ces dernières n'ont pas de but lucratif. Cette contribution pourrait déséquilibrer leur modèle économique, menaçant ainsi leur forte contribution à l'accès aux soins des Français et à la promotion d'une complémentaire santé accessible pour tous. Par ailleurs, le calcul de cette contribution est fondé sur la baisse des dépenses de soins liée au confinement intervenu de mars à mai 2020. Cet amendement vise donc à garantir une meilleure transparence et une plus grande cohérence de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d'assurance maladie en utilisant comme référence les cotisations perçues en 2020.

sans étude préalable, notamment sur le rattrapage de la consommation de soins. Par conséquent, il est proposé de créer un dispositif réglementaire plus souple

Je comprends votre argumentation et les craintes que vous exprimez. Toutefois, l'adoption de ces amendements aboutirait à taxer deux fois- en 2020 et en 2021 -le montant des primes et des cotisations.

que les complémentaires peuvent tout à fait assumer.

de covid-19. Ainsi présentée, la mesure risque de toucher directement les comptes des régimes collectifs complémentaires pilotés par les branches professionnelles et hébergés par des organismes assureurs recommandés. Les organismes assureurs seront ainsi tentés de répercuter cette contribution sur les régimes collectifs de branche en relevant à due concurrence les cotisations patronales et salariales. Or ces régimes sont déjà souvent tout juste à l'équilibre, sinon en déficit. D'une part, l'augmentation des cotisations salariales et patronales est tout à fait inopportune en période de crise économique. En effet, les entreprises sont déjà fortement fragilisées, particulièrement les TPE-PME, qui sont les principales souscriptrices souscriptrices des contrats collectifs de branche organisant une mutualisation. D'autre part, cette augmentation risque de dissuader les entreprises de rejoindre les régimes de branche, et donc de réduire la mutualisation qu'ils doivent en principe favoriser, particulièrement en période de crise sanitaire. Il est donc proposé que la contribution exceptionnelle ne puisse pas être répercutée sur les régimes collectifs complémentaires de branche gérés par les organismes recommandés.

elle bénéficie d'une exonération de contribution patronale de 20 % sur la valeur des actions attribuées au jour de l'attribution, à condition qu'au jour de la décision d'attribution, elle n'ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L'exonération de contribution patronale s'applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. Le présent amendement vise à étendre l'exonération de cotisations patronales aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire (ETI), au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776

et les dirigeants. Par conséquent, l'extension de l'exonération existante pour les PME aux ETI permettrait un développement croissant de ces dispositifs et irait dans le bon sens.

l'actionnariat salarié. Dans le document transmis aux organisations syndicales et patronales, le ministère se fixe comme objectif de mieux lier la rémunération du travail à la performance de l'entreprise, qu'elle soit économique ou sociale. À cette fin, il propose la création de dispositifs de rémunération variable collective simplifiés pour les petites entreprises. Il propose en outre le développement de l'actionnariat salarié, par exemple en distribuant une part d'actions gratuites aux salariés au titre de la participation, ou en renforçant l'incitation au versement d'épargne salariale dans les fonds d'actionnariat salarié.

pas l'actionnariat des entreprises. La crise économique de 2020 n'est que l'ultime soubresaut de l'économie capitaliste. Plutôt que de développer les actions gratuites, ce qui aura pour effet d'assécher davantage les recettes de la sécurité sociale,

Par cet amendement, nous souhaitons en finir avec la désocialisation des heures supplémentaires instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2019, renforcée par les mesures d'urgence économique et sociale

la nécessaire réduction du temps de travail, la désocialisation des heures supplémentaires incite les salariés à travailler davantage. La rengaine du « travailler plus » est un non-sens. Elle ne favorise ni la création d'emplois

le dispositif actuel ne reprend que partiellement le dispositif en vigueur entre 2007 et 2012, qui avait prouvé son efficacité. Dans le contexte de la crise sanitaire et compte tenu de la nécessité de relancer l'économie, il est proposé d'étendre ce dispositif en supprimant l'ensemble des cotisations afin de le rendre plus incitatif.

une incitation aux heures supplémentaires une exonération de cotisations. Il ne me paraît pas davantage opportun de supprimer une mesure de pouvoir d'achat, c'est-à-dire une exonération de cotisations salariales,

Mise en place par le Gouvernement, cette mesure, qui s'ajoute à l'exonération d'impôt sur le revenu, a permis un gain de pouvoir d'achat annuel de 455 euros en moyenne pour les salariés effectuant des heures supplémentaires, ce qui est considérable. Pour les cotisations patronales, une déduction forfaitaire de 1,5 euro par heure supplémentaire effectuée existe déjà pour les entreprises de moins de vingt salariés, pour lesquelles il est nécessaire de favoriser la souplesse dans l'organisation du travail. Une extension de cette déduction à l'ensemble des employeurs aurait, dans le contexte actuel, un effet assez faible, voire nul, sur le nombre d'heures supplémentaires effectué. En revanche, elle aurait un coût très important pour les finances publiques. Dans le contexte actuel, le Gouvernement préfère donc concentrer ses efforts sur le soutien aux entreprises dans les secteurs les plus affectés

Pour des raisons idéologiques, on a fait croire que c'était le coût du travail qui pénalisait la compétitivité en France. La sécurité sociale n'a pas à se substituer aux

pour accroître davantage la rentabilité du capital.

On oublie d'expliquer que les cotisations sociales sont du salaire différé, et que c'est bien plus important pour les bas salaires que pour les hauts salaires. Le salaire différé signifie aussi une protection sociale et des droits à la retraite accrus. C'est également une protection supplémentaire pour les hauts salaires. Il faudrait cesser de toujours parler des cotisations sociales comme étant des charges.

L'article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales avait, dans le but de soutenir le pouvoir d'achat des ménages, ouvert aux employeurs la possibilité de verser à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à trois SMIC une prime exonérée, dans la limite de 1 000 euros, d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle et de tout autres cotisation et contribution dues. L'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 a reconduit cette prime en la subordonnant à l'existence d'un accord d'intéressement. Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ont été assouplies par l'ordonnance n° 2020-385 du 1 avril 2020 en vigueur depuis le 2 avril 2020. L'ordonnance du 1 avril 2020 a supprimé la condition de l'existence d'un accord d'intéressement, de sorte que cette prime peut désormais être versée par tous les employeurs. Elle a également, sous certaines conditions, fixé à 2 000 euros le montant maximum de prime bénéficiant des exonérations fiscales et sociales. sociales. Cet amendement vise à prévoir que le principe, les exonérations, ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1 janvier 2021, selon les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-385 du 1 avril 2020.

concluant un accord d'intéressement ou en donnant la possibilité aux plus petites entreprises de mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale de l'employeur ou encore d'appliquer directement un accord d'intéressement négocié au niveau de la branche. Cet effort en faveur du partage de la valeur se poursuit avec la suppression du forfait social sur l'abondement employeur, qui correspond à un versement volontaire du salarié dans le cadre de l'actionnariat salarié. C'est d'ailleurs

afin de répondre à l'urgence et de permettre à tous les employeurs de récompenser rapidement les salariés particulièrement mobilisés durant la crise sanitaire. En proposant seulement de pérenniser l'exonération des primes, on ne favorise pas

Cependant, la baisse des dépenses constatée pour ce premier semestre 2020 serait de 30 millions d'euros pour la Camieg et de 35 millions d'euros pour la CPRP SNCF.

et ne correspondent pas à la réalité comptable. Avec cet amendement, nous demandons au Gouvernement de revoir le montant de la contribution demandée à ces deux caisses.

soit 1 200 euros par ayant droit, ce qui est un effort considérable pour les salariés et les retraités des industries électriques et gazières.

du Gouvernement ? En complément des informations données par le rapporteur général, je rappelle que, depuis sa création en 2007, la Camieg dégage des excédents importants sur les fonds d'assurance maladie complémentaire obligatoire qu'elle gère. Le montant de ses réserves s'élèvera à 458 millions d'euros en 2021, et à 1 milliard d'euros en 2035. Vous le savez, la crise sanitaire a entraîné une baisse des dépenses des régimes complémentaires, en écho à la forte mobilisation de l'assurance maladie obligatoire de base pour lutter contre le virus. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a lancé une concertation avec l'ensemble des employeurs

vous en donner quelques détails : le Gouvernement s'est engagé à procéder, dès le 1janvier 2021, à une baisse des cotisations pesant sur les assurés et les retraités. Par exemple, pour un salaire brut mensuel de 2 500 euros, la baisse des cotisations sera d'environ 11 euros par mois, soit une baisse annuelle de 132 euros. Le Gouvernement procédera également à une amélioration de la prise en charge des frais d'optique de ces assurés. En conclusion, ces mesures visent ici un double objectif : elles participent, d'une part, à la relance et à l'amélioration directe du pouvoir d'achat des salariés et des pensionnés des industries électriques et gazières

afin de permettre à chacun de participer aux commémorations du 11 novembre, et en accord avec la commission et le Gouvernement, nous lèverons notre séance vers dix-huit heures.

Cette somme est censée compenser les déséquilibres des autres caisses de l'assurance maladie. Alors que le Gouvernement appelle à l'équilibre des comptes sociaux, il est incompréhensible

qui gère les prestations maladie et maternité pour le régime général, mais aussi l'assurance maladie complémentaire de ses assurés, dégage des excédents importants depuis sa création en 2007.

des réserves de la Camieg ! Les fédérations syndicales des industries électriques et gazières nous ont contactés pour nous faire part du caractère disproportionné, injuste et incompréhensible de cette

Les électriciens et gaziers font partie des salariés qui étaient en première ligne lors de la pandémie. Les excédents de la caisse doivent servir à améliorer leurs droits en matière de protection sociale. La commission des affaires sociales ayant émis

Ce plafond est une valeur de référence, indexée sur le salaire moyen par tête, et utilisée pour le calcul des cotisations et des prestations. On peut comprendre intuitivement que sa diminution, résultant d'une baisse artificielle des salaires nominaux, liée à la crise sanitaire et notamment au chômage partiel, pourrait effectivement poser problème. le fait de fixer un plafond pour 2021 équivalent à celui de 2020, pour neutraliser les effets du chômage partiel, aura des effets très concrets sur les cotisations et sur les prestations plafonnées et, donc, sur les assurés. Or vous ne proposez pas d'estimation complète de ces effets

Avez-vous, madame la secrétaire d'État, des éléments chiffrés supplémentaires à nous communiquer sur les conséquences de cette modification du plafond, sur les différentes déformations conjoncturelles en résultant, par exemple sur les niveaux de prestations en espèces, en somme, sur la réalité des assurés ? L'amendement

Si l'on comprend bien la nécessité d'une adaptation circonstancielle de la méthode de calcul actuelle, du fait de la crise économique et sociale et des conséquences du recours au temps partiel, il reste en réalité que rien ne justifie une modification pérenne du dispositif actuel, et ce d'autant moins que, de l'aveu même du Gouvernement, une modification réglementaire était possible à la lecture de l'étude d'impact. nous considérons donc que la représentation nationale n'a pas été correctement informée par le Gouvernement des raisons pour lesquelles cette réforme systémique, présentée comme anecdotique, doit devenir pérenne, et de ses conséquences réelles sur les finances des organismes de protection sociale, les exonérations de cotisations sociales et les niveaux de prestations en espèces. Quel est l'avis de la commission ? La commission-

avant la crise très singulière que nous traversons. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que les textes juridiques en vigueur ne prévoient rien pour éviter cet effet. Le montant du PASS, vous le savez, n'a jamais diminué depuis sa création. Jamais

de rendre pérenne la modification du mode d'évolution du plafond, elle répond ici aux besoins de sécurisation juridique des entreprises, mais aussi des assurés. Si nous n'acceptons pas cette baisse pour les droits sociaux acquis en 2021, pourquoi l'accepterions-nous pour les années suivantes ? En l'occurrence, la mesure

La parole est à M. Jean-Luc Fichet, sur l'article. Le dispositif d'exonération applicable pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi (TO-DE) permet aux employeurs qui embauchent des travailleurs saisonniers de bénéficier d'une exonération de cotisations patronales.

De nombreux secteurs agricoles ont en effet été particulièrement affectés par l'épidémie de la covid-19 du fait de leur dépendance au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, dont l'activité a été et se retrouve à nouveau interrompue par les mesures d'interdiction d'accueil du public. Si cette prorogation va dans le bon sens, elle nous paraît néanmoins insuffisante au regard des conséquences économiques exceptionnelles de la crise. En outre, au-delà de la situation actuelle, cette exonération se justifiait déjà par la difficulté à laquelle les producteurs agricoles sont confrontés pour recruter des travailleurs saisonniers, notamment du fait de la concurrence des pays européens. La suppression du travail occasionnel représenterait ainsi une augmentation de charges de 189 euros par saisonnier et par mois pour les 900 000 contrats concernés. En année pleine, ce sont environ 70 000 entreprises qui bénéficient actuellement de ce dispositif, soit près de la moitié des entreprises du secteur de la production agricole employant des salariés.

Il nous faut donc envoyer un signal fort, en pérennisant ce dispositif d'exonération. Ainsi, nous donnerons à nos producteurs les moyens de continuer à employer de la main-d'oeuvre locale. Le premier confinement a révélé l'engouement des Français pour les produits de nos agriculteurs. Mais, sans le dispositif TO-DE, ces derniers devront faire appel à des travailleurs de l'étranger pour assurer leur production et les produits français ne pourront pas rivaliser avec ceux de nos concurrents. Nos agriculteurs sont d'accord pour se moderniser et mieux respecter chaque jour les normes environnementales. Encore faut-il qu'ils soient soutenus et accompagnés durablement ! Nos agriculteurs ont besoin de visibilité.

rectificative, il a mis en place des exonérations afin de soutenir les secteurs agricoles les plus durement affectés par les conséquences économiques des mesures prises pendant l'état d'urgence sanitaire, en particulier les activités qui étaient très directement dépendantes des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration-

l'emploi saisonnier agricole n'a pas été massivement affecté par la crise. Le volume d'embauches de travailleurs occasionnels bénéficiant de cette exonération est même en légère progression au cours du premier semestre. À la fin du mois de juin, il était de 4,7 % supérieur à celui de l'année précédente à la même période. La reconduction à titre provisoire de cette exonération particulière jusqu'au 31 décembre 2022 représente une mesure de soutien supplémentaire de 130 millions d'euros par an, pour certaines filières agricoles ayant recours à l'emploi saisonnier.

pour présenter l'amendement n° 693 rectifié . L'embauche d'un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Ce dispositif, qui devait être supprimé au 1 janvier 2021, va néanmoins perdurer jusqu'au 1 janvier 2023, comme le prévoit l'article 13 du présent PLFSS. Toutefois, il est limité aux agriculteurs employeurs de main-d'oeuvre à titre individuel ou collectif- en commun. Cet amendement vise à inclure les 12 000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main-d'oeuvre auxquelles les exploitants agricoles délèguent des travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole, ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l'exonération. Exclues depuis la loi de finances 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d'un coup de pouce fiscal de 15 millions d'euros,

exclues depuis 2015 du champ d'application du dispositif TO-DE, car elles disposent d'une clientèle diversifiée et sont ainsi moins soumises à la saisonnalité que les exploitations agricoles. Par construction, leur personnel est plus qualifié. En pratique, exonérer ces entreprises aurait pour effet de les inciter à recourir à des contrats saisonniers, alors même que leur activité justifie plutôt le recours à des salariés permanents. La différence de situation dans laquelle se trouvent les Etarf par rapport aux exploitations agricoles, ainsi que la volonté du Gouvernement de lutter contre la précarisation des emplois dans ce secteur, justifie leur exclusion du dispositif TO-DE. Je vous rappelle que ces entreprises bénéficient

prévoit le versement d'une indemnité de précarité au-delà des exigences légales. Actuellement, l'indemnité conventionnelle est prise en compte dans le calcul et conduit mécaniquement au dépassement du seuil de 1,2 SMIC au-delà duquel l'exonération diminue. Dans la période actuelle, ces dispositions conventionnelles favorisant le pouvoir d'achat des travailleurs saisonniers ne doivent pas se retourner contre les employeurs, en leur faisant perdre une partie des exonérations auxquels ils auraient droit s'ils ne versaient pas cette indemnité.

est à Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous souhaitons que les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique soient assujetties aux cotisations et contributions sociales. Ce nouveau dispositif de non-assujettissement, couplé

le bas ! Les protections attachées au statut de la fonction publique devraient, au contraire, faire davantage figure d'exemples en termes de droits au travail. Le dispositif de rupture conventionnelle ainsi importé dans la fonction publique est d'ailleurs un nouvel outil des employeurs

? L'avis est défavorable. Même si la commission ne s'enthousiasme pas face à des exonérations de CSG, cela peut davantage se justifier au moment où une personne perd son emploi. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les précédents votes du Sénat en la matière.

1,7 point. La conséquence fut évidemment une perte de pouvoir d'achat pour les retraités et les fonctionnaires. Selon le rapport annuel sur l'état de la fonction publique pour l'année 2019, le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique territoriale a baissé, en moyenne, de 0,4 %. Nous proposons de revenir sur cette mesure, complètement injuste, en supprimant la hausse de la CSG

nos concitoyens. Si l'on veut relancer l'économie, il faut redonner du pouvoir d'achat et revenir à une plus grande solidarité entre le capital et le travail !

en 2018 et 2019. Enfin, et pour terminer, une hausse du taux de CSG sur les revenus du capital est à exclure dans un contexte où le Gouvernement- je le redis avec force -s'est engagé à ne pas augmenter

J'entends bien, messieurs, l'argument selon lequel il faut favoriser l'installation des jeunes en agriculture. J'y suis tout à fait favorable et je pense que la commission partage aussi ce sentiment. Vous considérez que

ayant eux-mêmes largement communiqué sur la généralisation de cette médiation. Une rubrique thématique à destination des cotisants est disponible sur le site internet des Urssaf. La saisine du médiateur peut d'ailleurs se faire directement en ligne sur ce site en remplissant un simple formulaire. Il est très important que la médiation reste utilisée à bon escient, dans les cas où elle est véritablement nécessaire. Pour mémoire- et je ne doute pas que vous le sachiez la médiation vise à apporter une réponse amiable rapide à des situations spécifiques pour lesquelles les dispositifs existants de règlement des différends se révèlent inadaptés. Introduire cette information sur toute réclamation ne me semble pas approprié pour favoriser le dialogue : les agents des organismes doivent rester les principaux interlocuteurs des cotisants et traiter les questions qu'ils peuvent résoudre. Ces réclamations doivent pouvoir suivre un cours normal. Ce n'est vraiment qu'en cas de blocage ou de rupture du dialogue, ce qui peut aussi arriver,

Cette différence de traitement est évidemment inéquitable, en particulier à l'égard des établissements publics, qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes ; il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l'aide sociale, les Ehpad publics sont en première ligne, on le sait, pour assurer l'accessibilité à ces établissements des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs d'hébergement inférieurs en moyenne de 500 euros par mois à ceux du secteur commercial. les tarifs d'hébergement n'ont pas suivi l'évolution des charges et leur augmentation est, depuis bientôt dix ans, systématiquement inférieure à l'inflation, ce qui a rendu impossible pour beaucoup d'Ehpad publics le maintien d'une capacité d'autofinancement suffisante.

sociale. En revanche, dans ce contexte financier, il ne convient pas de créer de nouveaux dispositifs d'exonération pérennes. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable

Elles ont également joué un rôle crucial dans les services essentiels tels que la production alimentaire et la chaîne d'approvisionnement, les secteurs du nettoyage et de la blanchisserie, ainsi que celui des soins. Les femmes sont également surreprésentées dans les secteurs qui ont été parmi les plus durement touchés par les mesures de lutte contre la covid-19 : l'accueil, la vente au détail, les loisirs, les librairies, etc. En outre, l'inégalité préexistante entre les sexes- par exemple les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes -et les déséquilibres flagrants dans la répartition par sexe des soins non rémunérés et du travail domestique sont susceptibles d'amener les femmes à renoncer à participer au marché du travail pendant la pandémie et au-delà. Les quarantaines, les fermetures d'écoles et d'autres restrictions de mouvements visant à freiner la propagation de la covid-19 ont contribué à la forte augmentation de la violence fondée sur le genre, en particulier la violence domestique au sein des couples. Face à l'accroissement des inégalités salariales durant la covid-19, et malgré l'inscription dans la loi du principe d'égalité salariale depuis 1972, il faut envoyer un signal

celui d'augmenter le coût du travail, ce qui n'est, selon nous, pas souhaitable. L'employeur pourrait être amené à absorber cette hausse par différents moyens, par exemple- c'est possible -en substituant à des CDI à temps

la question de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes par les employeurs. Je précise à cet égard que des moyens existent aujourd'hui pour sanctionner les comportements les moins vertueux, notamment la pénalité prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail,

indûment versées se prescrit sur trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. En résumé, l'Urssaf peut réclamer aux cotisants des sommes sur une période plus longue que le délai auquel elle est elle-même soumise en cas de remboursement.

Vous justifiez cette demande par la différence qui existe entre la période pendant laquelle ce remboursement peut être demandé- trois années depuis que la somme payée est exigible -et celle pendant laquelle l'Urssaf peut réaliser un redressement- les trois années civiles précédant l'année en cours. En réalité, cette différence s'explique le moment essentiel pour faire courir le délai de prescription est celui de la connaissance d'un droit. Par ailleurs, la connaissance par le cotisant du droit à demander le remboursement d'un indu part nécessairement à compter du jour où il paie ses cotisations. Aussi, les trois années sont décomptées à partir de cette date. En revanche, l'Urssaf ne peut détecter une anomalie dans les cotisations versées qu'à l'occasion d'un contrôle. Or les contrôles sont réalisés uniquement sur une année civile entière. Les Urssaf ne contrôlent donc que les années antérieures à l'année au cours de laquelle le contrôle est réalisé. Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur cet

fonction d'interlocuteur, lequel pourrait être saisi par le cotisant en cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification. Aujourd'hui, en cas de contrôle, le cotisant est seul face à l'inspecteur. Il serait donc judicieux de pouvoir avoir recours à un tiers

est défavorable, monsieur Chasseing. La durée d'un contrôle dépend plus de la complexité d'un dossier que de la taille de l'entreprise. Une telle disposition risque de constituer une incitation forte à laisser traîner les choses. Quel est l'avis du Gouvernement

Je rappelle que les procédures de contrôle sont encadrées par un formalisme destiné à sécuriser les relations entre l'entreprise et l'organisme de recouvrement lors de la procédure. Le législateur a admis la limitation de la période de contrôle de l'Urssaf pour les entreprises de moins de 10 salariés à trois renouvelables une fois- donc six mois. Ce dispositif a été étendu par la loi Essoc aux entreprises de moins de 20 salariés à titre expérimental pour trois ans. Une autre expérimentation, également pour une durée de trois ans, limite à neuf mois les contrôles réalisés dans les entreprises de moins de 250 salariés, toutes administrations

dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Le donneur d'ordre est tenu de vérifier, lors de la conclusion d'un contrat portant sur une obligation d'une certaine valeur, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, À défaut de procéder à ces vérifications, et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d'ordre peut être poursuivi pénalement et devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant. Il peut également perdre le bénéfice des exonérations et des réductions de cotisations applicables à ses salariés sur toute la période où le délit de travail dissimulé du sous-traitant constaté. À l'heure où les Urssaf montrent qu'elles entendent privilégier le dialogue avec les cotisants, le système devrait être revu. Il convient donc d'inscrire dans la loi que l'absence de délivrance de l'attestation de vigilance ne peut intervenir qu'au terme de la procédure contradictoire.

car l'entreprise ne disposera pas davantage de l'attestation de vigilance pendant une période d'attente qu'après un refus. Quel

été faite plusieurs fois. Vous demandez, lorsqu'un contrôle a conduit à révéler une fraude, que l'on attende la fin du délai d'échange contradictoire pour retirer à une entreprise son attestation de comptes à jour délivrée par les Urssaf pour candidater à des marchés publics ou privés. En d'autres termes, un cotisant qui a réalisé un travail dissimulé

de continuer à obtenir un quitus utilisable après sa verbalisation, ce qui n'est pas l'objectif du Gouvernement. Je ne peux donc qu'être défavorable à votre amendement. Je le retire,

ses observations et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure. Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximale de trois mois.

n° 212 rectifié. En 2018, près de 4 millions de Français résidaient dans une zone sous-dotée en médecins généralistes. Ce problème touche aussi bien les territoires ruraux et ultramarins que certaines grandes agglomérations. En Île-de-France en particulier, on constate une baisse inquiétante du nombre de praticiens libéraux depuis plusieurs années. En dix ans, la région a perdu 2 000 médecins généralistes. Dans certaines communes, il faut attendre de nombreux mois pour obtenir un rendez-vous. selon le président de l'Union régionale des professionnels de santé, l'URPS, 48 % des médecins libéraux franciliens ont plus de 60 ans et sont susceptibles de partir à la retraite dans les cinq prochaines années. Dans ce contexte, de nombreux médecins continuent à travailler après l'âge légal, notamment parce qu'ils refusent d'abandonner leur patientèle. Nous proposons d'encourager cette démarche en instituant un abaissement de charges sociales pour les médecins qui font ce choix dans les zones les moins bien dotées.

madame la ministre,

Ainsi, les praticiens retraités exerçant dans ces territoires sont exonérés de cotisations au régime des prestations complémentaires de vieillesse sur les 80 000 premiers euros de revenus.

un effort financier annuel de l'ordre de 36 millions d'euros. Elle bénéficie à un peu plus de 44 000 nouveaux agriculteurs, qui acquittent déjà de très faibles montants de cotisations sociales de début d'activité.

dès lors que le journaliste exerce à l'étranger. Elles s'affranchissent donc des cotisations sociales que le contrat de travail implique. Cet amendement, que je présente au nom de mon groupe, vise à affirmer la nature du contrat

presse française. Il tend à modifier la disposition du code du travail relative à la présomption de salariat dont bénéficient tous les journalistes professionnels, y compris les pigistes, depuis la loi Brachard de 1935 et la loi Cressard de 1974. est de conforter l'application du droit du travail et du droit de la sécurité sociale français aux journalistes salariés d'entreprises de presse françaises qui effectuent une mission à l'étranger. Comme les signataires de cet amendement,

tant par la législation nationale, avec l'article L. 7111-3 du code du travail, que par la législation européenne, avec le règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome

Le versement des cotisations, en France ou dans l'État du lieu d'exécution de la prestation, dépend du statut du journaliste et de l'existence, ou non, d'une convention bilatérale de sécurité sociale. À défaut, la protection sociale du journaliste exerçant à l'étranger peut être assurée par le versement de cotisations volontaires à la caisse des Français de l'étranger.

instaure une exonération de la part patronale des cotisations sociales des salariés des exploitations et entreprises du secteur de la vigne ayant connu, en 2020, une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 20 % par rapport à l'année précédente.

Les mesures prises pour endiguer la propagation de la pandémie, au demeurant nécessaires, emportent des conséquences dévastatrices pour la filière brassicole depuis mars dernier, compte tenu de la grande dépendance de celle-ci aux secteurs des cafés, hôtels et restaurants. Comme d'autres secteurs, les 2 000 brasseries, dont 98 % de PME et de TPE, réparties sur tout le territoire métropolitain et ultramarin, ainsi que l'ensemble de la filière brassicole, font face à de lourdes pertes qui vont se prolonger et s'aggraver avec le reconfinement décidé par le Gouvernement et les sombres perspectives à venir.

Les dispositifs de soutien indispensables mis en place par l'État depuis le début de cette crise sont insuffisants pour permettre à ces jeunes entreprises de maintenir leur activité dans les prochains mois, alors que s'ouvre une période qui sera décisive pour la survie de la filière. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour

plus de 5 milliards d'euros, d'après les prévisions. Les activités de fabrication de bière bénéficient déjà directement de ces exonérations. L'article 6 crée de nouvelles mesures analogues qui concerneront également la filière brassicole. L'exonération de cotisations sociales et l'aide au paiement des cotisations, dont bénéficient les employeurs, ainsi que les mesures de réduction applicables aux non-salariés, s'ajoutent à d'autres dispositifs de soutien spécifiques comme la prolongation du Fonds de solidarité ou la prise en charge à 100 % du chômage partiel, sans même citer le dispositif fiscal. Ces amendements visent à établir l'exonération de cotisations sociales pour les employeurs agricoles travaillant dans le secteur de la fabrication de bière, selon le niveau de perte de chiffre d'affaires en 2020.

Par ailleurs, pour la filière brassicole, une mesure exceptionnelle d'indemnisation forfaitaire visant à compenser une partie des préjudices causés par les pertes de débouchés sera financée à hauteur de

cidre, le pommeau et autres produits de Normandie. Même motif, même punition : perte de chiffre d'affaires, difficultés,

Cet amendement vise à réparer une injustice historique et à aligner les droits de mutation et de circulation des vins produits en méthode ancestrale, titrant moins de 7,5 degrés d'alcool, sur ceux qui s'appliquent aux vins pétillants peu alcoolisés. Ainsi, le tarif par hectolitre passerait de 9,59 euros

pour les vins titrant à moins de 8,5 degrés d'alcool, notamment les pays de l'Europe du Nord, la Belgique et le Royaume-Uni. Le degré d'alcool des vins en méthode ancestrale est en moyenne de 7,5 degrés, mais ces breuvages sont pourtant classés aujourd'hui dans la même catégorie que les vins mousseux en méthode dite traditionnelle, lesquels titrent entre 10 et 12 degrés en moyenne. réparer cette anomalie en alignant les droits de circulation de ces vins sur ceux du cidre, du poiré, de l'hydromel et des jus de raisin légèrement fermentés, soit 1,36 euro

Aujourd'hui, nous vous proposons, par cet amendement visant expressément la clairette de Die, d'aligner, à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2022, les droits de circulation frappant ce vin effervescent qui s'appliquent aux vins pétillants peu alcoolisés. On passerait ainsi d'un tarif de 9,59 euros l'hectolitre à 1,36 euro jusqu'au 31 décembre 2022. Cet amendement vise à sauver la filière viticole du secteur de Die et du Diois, qui rencontre actuellement de graves difficultés économiques. Plus qu'une filière agricole, la production de clairette de Die constitue l'activité économique principale de la vallée du Diois, ce qui en fait, au-delà du produit, un symbole et un atout de l'attractivité du territoire.

Cette proposition ne repose sur aucune justification au regard des impératifs de santé publique ou de considérations économiques. Cette réduction de taxes, au demeurant, ne ferait qu'accroître

de Die. Il est inenvisageable et, surtout, juridiquement impossible de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques à l'égard de tous les autres producteurs de vins mousseux, même à titre temporaire. Par ailleurs, je rappelle que le Gouvernement a déjà engagé un plan de soutien à la filière viticole de 250 millions d'euros. Pour toutes ces raisons, et malgré le charme de la clairette de Die, l'avis est défavorable. La parole

devenir nettement moins consensuels. En cette période de crise, il est sage de s'en tenir aux dispositifs présentés par le Gouvernement, qui seront améliorés par notre assemblée au cours des débats, grâce à nos propositions. C'est la raison pour laquelle je vous invite à rejeter l'ensemble de ces amendements. La parole

la mi-octobre, avec 70 % d'avances pour les aides découplées et 85 % pour l'indemnité compensatoire de handicap naturel. Le solde leur sera versé d'ici à la mi-décembre. la mi-décembre. Ils bénéficieront, en outre, de dégrèvements de taxe sur le foncier non bâti. Votre amendement conduirait à calculer les cotisations au titre de 2020 en fonction des seuls revenus de cette même année, ce qui pourrait être favorable en termes de moindre cotisation si ces assurés ont connu, cette année-là, une baisse importante de leurs revenus. Cependant, le calcul qui minore les cotisations minorerait également les droits sociaux correspondants, notamment en matière de retraite. Il n'est pas souhaitable, par ailleurs, de modifier les règles relatives à l'assiette des prélèvements dès qu'une crise réduit les revenus et d'abandonner, chaque fois, le recouvrement des cotisations dues au titre des années antérieures. Cela ne constitue pas une solution viable viable sur le long terme. J'ajoute que le mécanisme de calcul qui consiste à retenir pour assiette les revenus des trois dernières années n'est pas adapté à des revenus variables, puisqu'il conduit à un écart important entre l'année lors de laquelle le revenu est perçu et celle

ce travail doit être entrepris, mais de façon plus structurée que par le biais d'un amendement. Vous le savez, il est impossible de faire coexister deux dispositifs- une assiette triennale et une assiette contemporaine -entre lesquels on pourrait choisir d'une année à l'autre.